Monsieur le président,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

M. le président du Sénat a été informé, par lettre en date du 16 avril 2018 de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, que, à la suite de l'annulation, le 13 avril 2018, de l'élection de M. Sébastien Leroux, sénateur de l'Orne, le siège, devenu vacant à compter du 14 avril 2018 à zéro heure, sera pourvu, selon les termes de l'article L.O. 322 du code électoral, par une élection partielle organisée à cet effet dans un délai de trois mois. Mes chers collègues, par lettre en date du lundi 16 avril 2018, le Gouvernement a demandé de compléter l'ordre du jour du jeudi 19 avril par l'inscription de la suite éventuelle de la proposition de loi de transposition de la directive du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. Acte est donné de cette demande. J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein :- d'une part, de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ;- d'autre part, de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur le projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen.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 adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis la loi Chevènement de 1999 et sous tous les gouvernements, quelle que soit la majorité au pouvoir, l'intercommunalité s'est développée et transformée dans notre pays.

territoriale de la République, la loi NOTRe, a élevé le seuil des intercommunalités à 15 000 habitants, hors dérogation, pour des raisons de densité de population. Sur le plan fiscal, la suppression de la taxe professionnelle en 2010 a engendré de nouvelles recompositions, mais là n'est pas le sujet aujourd'hui- nous réétudierons prochainement la question de la refonte de la fiscalité locale. Enfin, sur le plan des compétences, la loi NOTRe a procédé à la répartition entre les différents niveaux de collectivités pour répondre à trois objectifs : la lisibilité pour le citoyen, l'efficacité des politiques publiques et l'efficience économique. C'est le sujet dont nous débattons aujourd'hui en ce qui concerne l'eau et l'assainissement. Après avoir été longtemps une compétence facultative, puis optionnelle,

la qualité de l'eau, l'accès à la ressource en eau et le portage des investissements est souvent débattue, et les enjeux qui nous attendent, collectivement, en matière de qualité et de ressource en eau sont colossaux. questionner sur l'efficience de nos dispositifs et le portage de nos investissements. Du point de vue de l'accès à l'eau, l'impératif écologique ne cesse de se rappeler de se rappeler à nous, avec des épisodes de sécheresse de plus en plus longs. La topographie, la géographie et la fragmentation des réseaux ont dessiné des situations très disparates En matière de qualité de l'eau, les derniers épisodes d'inondation ou de fortes pluies ont, par exemple, entraîné une pollution des eaux contenues dans les nappes phréatiques ou dans les zones de stockage, en zone urbanisée ou en zone non urbanisée, car les eaux pluviales se chargent en pollution tout au long de leur parcours. L'évolution de nos modes d'agriculture rend aussi nécessaire de repenser l'accès à l'eau et ses usages pour l'agriculteur. D'un point de vue économique, nos installations sont, en de trop nombreux endroits, vieillissantes ou vétustes. Les taux de fuite de nos réseaux avoisinent 30 % et atteignent parfois plus de 50 %. Ce sont ainsi plus de 1 milliard de litres d'eau qui sont captés, transportés, traités dans nos usines chaque année, mais qui n'arrivent jamais jusqu'au robinet. Pour répondre à ces enjeux et devant ces phénomènes grandissants,

Les communes ont également fait le choix de déléguer la compétence à des syndicats. Lors de mes nombreux déplacements, j'ai pu constater les situations très diverses, avec des syndicats parfois tout à fait remarquables. Dans le département de la Vienne, par exemple, le syndicat Eaux de Vienne prend en charge les compétences « eau et assainissement » sur la quasi-intégralité du périmètre du département afin d'avoir une vision unifiée de la compétence et de proposer un tarif absolument identique dans toutes les communes. Les intercommunalités peuvent d'ailleurs recourir à des modes de gestion différents- délégations de service public, régies ou autres statuts juridiques -pour

Les communes ne feront efficacement face aux risques d'amoindrissement de la qualité et de la ressource en eau que si elles interconnectent leurs réseaux et si elles mutualisent leurs moyens à des échelles plus larges.

en cours de transmission, préconise de piloter cette question à une échelle cohérente. Dans les zones urbaines et denses, la gestion des eaux pluviales est intimement liée à l'assainissement, notamment dès lors que le réseau est unitaire. Dans les zones moins denses,

qui fournit un exemple concret de la gestion intégrée dans le cadre du contrat de rivière, une compétence GEMAPI. Ces enjeux environnementaux se doublent d'enjeux financiers très importants. Les investissements sont nécessaires et sont aujourd'hui évalués à 5 milliards d'euros. Chaque euro dépensé en matière d'eau et d'assainissement doit permettre de conduire au robinet le plus grand volume d'eau. C'est de cette manière que nous réduirons la facture pour les collectivités et pour les usagers. de dégager de nouvelles marges de manoeuvre, il convient, pour certains, de mutualiser les moyens et les compétences. C'est le choix qu'a déjà fait la moitié des communes en transférant cette compétence à l'intercommunalité.

Si vous le permettez, je vais terminer mon exposé ! Nous avons donc travaillé, disais-je, à trouver un texte de compromis qui concilie les enjeux d'un nécessaire transfert avec ceux, légitimes, d'une adaptation à certaines réalités locales. Tel est le sens de la mission que m'avait confiée le Premier ministre. Aussi ai-je décidé à l'automne dernier d'installer un groupe de travail comprenant seize parlementaires nommés par chaque président des deux chambres. Nous avons commencé les travaux le 7 novembre dernier et nous avons auditionné les associations d'élus du bloc local, ainsi que les principaux acteurs de l'eau, privés ou publics- comités de bassin, agences de l'eau, fédération des entreprises de l'eau et fédération des collectivités concédantes et régies.

Les réflexions et propositions du groupe de travail en matière d'eau et d'assainissement ont permis d'aboutir à un premier accord, qui a été présenté lors de la Conférence nationale des territoires du 14 décembre, à Cahors.

En synthèse de la réunion de Cahors, nous n'allons pas revenir, a dit le Premier ministre, sur le principe du transfert il n'y a rien à voir ! ... aux intercommunalités au 1 janvier 2020, qui nous paraît nécessaire pour mener à bien les travaux d'investissement dont les réseaux ont besoin. En revanche, nous avons admis la possibilité d'y déroger dans certaines circonstances jusqu'en 1926 ... Jusqu'en

Nous avons admis, disais-je, la possibilité d'y déroger dans certaines circonstances jusqu'en 2026 sur la base d'une minorité de blocage. Le groupe de travail s'est ensuite réuni le 19 décembre autour d'une proposition de texte,

dans l'examen de ce texte est donc assez simple, mesdames, messieurs les sénateurs : il s'en tiendra globalement à l'accord auquel est parvenu le groupe de travail, et c'est le sens de l'amendement de réécriture que nous avons déposé. d'un texte de compromis. Le groupe de travail a conclu sur une clause de sauvegarde des libertés communales en donnant la possibilité aux communes de s'opposer au transfert des compétences « eau » et « assainissement avant le 1 juillet 2019 si 25 % d'entre elles représentant au moins 20 % de la population s'expriment en ce sens. Cette possibilité est réservée aux communautés de communes, car, d'une part, ce sont elles qui couvrent majoritairement les zones de montagne et les zones rurales,

de travail a également souhaité introduire « un effet cliquet ». Ainsi, si des EPCI exercent déjà la compétence « eau » ou « assainissement au niveau intercommunal de manière facultative ou optionnelle, ils conservent leur exercice au niveau intercommunal, sans capacité de revenir en arrière. Il a aussi constaté que les vraies difficultés se concentraient sur l'eau et non sur l'assainissement. Ce constat nous a conduits à proposer

et se donner un délai supplémentaire la capacité de blocage que je viens d'évoquer pour transférer l'eau s'ils n'y sont pas prêts. Enfin, nous observons que la commission des lois du Sénat a fait sien l'article 3 relatif au mécanisme de représentation-substitution dans les syndicats, que j'avais tenu personnellement à intégrer,

Ainsi, entre ceux qui souhaitaient un transfert obligatoire et ceux qui souhaitaient un transfert optionnel, un compromis a été trouvé. Il est équilibré et raisonnable et permet de répondre aux attentes des acteurs pour une meilleure mise en oeuvre de ces compétences essentielles pour nos concitoyens. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, ... Encore heureux

Autrement dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières ! La parole Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le nous examinons aujourd'hui une proposition de loi de notre collègue député Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues, adoptée le 30 janvier dernier par l'Assemblée nationale, qui porte sur « la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes Le contexte, vous le connaissez, c'est celui de la loi NOTRe, avec le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération au 1 janvier 2020. Depuis, cette perspective de transfert a suscité, vous le savez tous, de fortes inquiétudes parmi les élus locaux. C'est d'ailleurs ce qu'avait parfaitement identifié la mission de contrôle et de suivi de la mise en oeuvre des dernières lois de réforme territoriale, que notre commission des lois avait mise en place en novembre 2015. en novembre 2015. Face à ces inquiétudes, le Sénat a adopté à l'unanimité, le 23 février dernier, la proposition de loi de nos collègues Bruno Retailleau et Philippe Bas, qui prévoyait le maintien de ces deux compétences dans le champ des compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération. Lors de son examen par l'Assemblée nationale, le 12 octobre 2017, et malgré le soutien du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Fabrice Brun, ainsi que de l'ensemble des groupes politiques, à l'exception du groupe majoritaire, cette proposition de loi a fait l'objet d'un renvoi en commission. Pourtant, comme au Sénat, les débats à l'Assemblée nationale avaient pointé les difficultés nombreuses et spécifiques rencontrées dans certains territoires. Je pense en particulier aux zones de montagne ou aux zones rurales, ou encore à celles dont le périmètre de l'intercommunalité ne permet pas d'envisager une gestion efficace à la suite du transfert de ces compétences à l'horizon 2020. Tout à fait ! Dans ce contexte et dans le cadre de la Conférence nationale des territoires, vous avez mis en place, madame la ministre, un groupe de travail composé de huit sénateurs et de huit députés, avec la charge, disiez-vous, de présenter des propositions consensuelles afin de répondre à ces difficultés. Ces travaux ont conduit au dépôt, puis à l'adoption de la proposition de loi de l'Assemblée nationale que nous sommes aujourd'hui appelés à examiner et qui se veut, si l'on vous en croit, la traduction législative de ces travaux. Pour autant, la logique sur laquelle repose cette proposition de loi est radicalement différente de celle du texte adopté par le Sénat le 23 février 2017. En effet, le Sénat proposait alors de maintenir l'eau et l'assainissement dans les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération, en laissant surtout aux élus locaux le soin de décider de l'opportunité d'un tel transfert et en donnant cette liberté au nom du principe de subsidiarité. L'Assemblée nationale, de son côté, a conservé le principe du transfert de ces deux compétences et concède simplement un aménagement de calendrier, et ce pour les seules communautés de communes. On peut d'ailleurs s'interroger et même nourrir quelques regrets, madame la ministre, pour votre penchant et pour ce choix de la proposition de loi de l'Assemblée nationale, de surcroît d'origine gouvernementale, plutôt que d'avoir opté en faveur de la proposition de loi sénatoriale

Ce n'est malheureusement pas le choix que vous avez retenu. Au demeurant, c'est regrettable et, plus encore, c'est dommageable, car, malheureusement, nous avons perdu beaucoup de temps, un temps précieux pour les collectivités locales Il n'y a pas lieu de revenir sur la proposition de loi que vous venez de présenter, madame la ministre : celle-ci n'a pas été jugée satisfaisante par notre commission des lois. D'abord, parce qu'elle maintient le caractère obligatoire du transfert et ne permet que d'obtenir un différé de cette obligation, en reportant celle-ci au plus tard au 1 janvier 2026, pour peu que soient réunies les conditions de minorité de blocage. À ce stade,

Car, en réalité, ce qui est proposé par ce texte est non pas une réelle minorité de blocage, mais un simple différé de calendrier ! Ensuite, parce que la proposition de loi concerne les seules communes membres de communautés de communes et non pas les communes membres de communautés d'agglomération.

qui ont des configurations parfaitement rurales : elles s'apparentent plus à des communautés de communes « rurales » qu'à de véritables communautés d'agglomération. il est difficile de comprendre qu'au motif que 70 % d'entre elles ont déjà bénéficié du transfert de ces deux compétences, rien ne devrait être fait pour les 30 % restantes, pour lesquelles ces transferts soulèvent, vous le savez, de véritables enjeux et des problèmes d'ordre technique et financier. Nous ne pouvons pas nous résoudre à suivre une telle marche forcée. Enfin, et cela n'est pas la moindre des craintes, parce que la gestion des eaux pluviales et celle des eaux de ruissellement dans les zones urbaines

la compétence « gestion des eaux pluviales », vous vous basez sur une jurisprudence du Conseil d'État de 2013. Or cette décision du Conseil d'État, madame la ministre, est antérieure à la loi NOTRe et ne permet donc pas d'apporter un éclairage suffisant et pertinent sur la portée des articles 64 et 66 Au demeurant, le cas d'espèce à l'origine de cette décision, qui concernait la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, visait un contexte particulier, celle-ci étant en effet dotée d'un réseau unifié de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.

puisqu'il l'attribuait à la compétence « eau et assainissement » dans sa globalité, en application du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur. plus, le service public de gestion des eaux pluviales urbaines est distinct de celui de l'assainissement, et les articles du code précité relatifs au service public de l'assainissement ne font référence qu'aux eaux usées et en aucun cas aux eaux pluviales. Enfin, madame la ministre, vous le savez, le rattachement de la gestion des eaux pluviales urbaines à l'assainissement soulève également de nombreuses difficultés techniques. Si, dans certains territoires, il existe une cohérence entre les réseaux d'assainissement et les réseaux d'eaux pluviales, dans d'autres, la gestion des eaux pluviales peut être plus efficacement assurée en lien avec d'autres compétences, comme la gestion de la voirie, laquelle peut d'ailleurs relever d'autres échelons. Quant au rattachement de la gestion des eaux de ruissellement à l'assainissement, il apparaît, lui aussi, totalement injustifié. Les difficultés que je viens de rappeler s'appliquent également à ce rattachement. nationale, sous couvert de précision et de coordination avec la jurisprudence du Conseil d'État, en a profité pour aller bien au-delà, puisque le Conseil d'État n'avait pas abordé cette question des eaux de ruissellement et ne s'était prononcé que sur les eaux pluviales. Et, madame la ministre, lors des débats que nous avons eus en décembre dernier sur l'exercice de la compétence GEMAPI, s'était interrogé à bon droit sur le rattachement de la gestion des eaux de ruissellement à la GEMAPI. C'est sur l'initiative de notre commission que nous avions finalement opté pour le financement d'actions y concourant par la taxe GEMAPI, mais la commission mixte paritaire n'avait pas retenu cette disposition. Le Gouvernement devait déposer un rapport au Parlement sur cette question en février dernier, ce qu'il n'a pas fait Bref, la question n'est toujours pas mûre, et pourtant on cherche à imposer d'office une solution qui n'est clairement pas satisfaisante. Voilà pourquoi, madame la ministre, la commission des lois a voté le rétablissement des principales dispositions de la proposition adoptée par le Sénat à l'unanimité en février 2017 qui prévoit le maintien des compétences « eau » et « assainissement » parmi les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération, ainsi que la sécabilité de la gestion des eaux pluviales au sein de la compétence « assainissement » de ces mêmes EPCI. ne faire aucune mention des eaux de ruissellement, cette dernière question ne pouvant être résolue sans disposer de l'ensemble des éléments nécessaires. De ce fait, seul le texte du Sénat permet, selon nous, de répondre exactement aux véritables attentes des communes concernées. Celles-ci ont besoin que le transfert de leurs compétences « eau » et « assainissement » aux intercommunalités soit rendu optionnel et que les conditions de ce transfert éventuel soient aménagées et assouplies.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,

aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération dès le 1 janvier 2020. Depuis, aucune commune, aucun territoire n'a perdu de temps

Il s'agit donc de répondre à cette légitime inquiétude des élus en assouplissant la loi NOTRe, et non de revenir en arrière, selon une posture que l'on pourrait qualifier de fausse défense des collectivités locales.

J'ai fait partie de ce groupe, et j'ai pu constater que l'ensemble des sensibilités y était représenté. Tous les participants avaient pour objectif de trouver un texte adapté à la réalité des enjeux, un texte de compromis. C'est à l'unanimité que les préconisations ont été remises. Celles-ci ont été reprises par le groupe Modem de l'Assemblée nationale, qui les a transformées en proposition de loi.

relatif à la gestion des eaux pluviales, mon groupe propose un amendement qui se veut également de compromis : il tend à ce que, pour les communautés de communes, la gestion des eaux pluviales demeure facultative, et, par conséquent, sécable de l'assainissement.

Une position équilibrée, pragmatique, dénuée de toute posture politique permettrait certainement de régler au bénéfice de nos collectivités la question des eaux pluviales qui les préoccupe. La parole est à M.

Monsieur le président, madame la ministre, les défenseurs des communes qui entendent les moderniser en les faisant disparaître dans des intercommunalités de plus en plus intégrées me rappellent l'ogre des contes il aimait tant les enfants qu'il les dévorait. Le malheur, c'est que, au terme d'une petite dizaine d'années de ces prétendues modernisations, ils auraient réussi, si la grande majorité des élus communaux n'avaient enfin réalisé quel marché de dupes, sous contraintes législatives et budgétaires, on leur proposait. Même les exécutifs des grandes intercommunalités, actifs militants jusque-là du transfert obligatoire à leur profit du maximum de compétences, constatent qu'en l'absence de financements nouveaux l'exercice a ses limites. La fausse proposition de loi, mais vrai projet de loi, dont nous débattons aujourd'hui, outre un repli politicien tactique, pourrait être le signe d'une hésitation des idéologues devant la réalité. S'il est en effet des compétences dont le bon exercice dépend des réalités physiques et humaines des territoires, des compétences pour lesquelles les regroupements artificiels seront financièrement calamiteux, ce sont bien celles de l'eau et de l'assainissement. Ici, la structure de gestion unique est bénéfique ; là, ce sont les regroupements partiels ; ailleurs, la gestion communale. Quand nos stratèges de bureau cesseront-ils de confondre la carte avec le territoire ?

domestiques, industrielles, voire les eaux résultant du lavage de la voirie par les précipitations habituelles, et la question, différente, du ruissellement calamiteux, source d'inondations, que l'on serait bien en peine de traiter. Comment peut-on dire sérieusement, comme notre chère ministre Jacqueline Gourault l'a fait, ici même, il y a quelques mois, que, si le ruissellement calamiteux « était rattaché à la compétence GEMAPI et non plus à la compétence " assainissement ", conformément à la jurisprudence de la Communauté européenne, cela poserait la question de la gestion des installations qui traitent à la fois les eaux usées et les eaux pluviales [ ...], et des stations d'épuration, qui relèvent logiquement de la responsabilité de la collectivité compétente au titre de l'assainissement

Autant dire que vous n'entendez rien faire ! Timide retour en grâce du principe de réalité, disais-je, que cette proposition de loi, ou rideau de fumée ? Reculer la date du transfert des compétences « eau » et « assainissement » à 2026 n'est pas revenir sur l'obligation du transfert de ces compétences prétendument siamoises.

précise qu'à tout moment jusqu'en 2026 l'exécutif des EPCI peut demander à vérifier si la minorité de blocage existe toujours. Si elle n'existe pas, quand les votes sont serrés, on pourra toujours lui donner un coup de pouce. Mais peut-être ai-je mauvais esprit

particulièrement celles qui rassemblent plusieurs bassins versants et celles qui sont en fait des communautés de communes de taille XXL. François Bonhomme et la commission des lois ont donc eu entièrement raison de disperser le rideau de fumée derrière lequel le Gouvernement tente de se cacher. Il faut que les choses soient claires et qu'elles soient dites, comme l'a fait notre commission : premièrement, le transfert aux EPCI, communautés d'agglomération ou de communes, des compétences « eau » et « assainissement » doit rester un choix des élus. Parfois, la raison l'impose, d'autres fois non. C'est ainsi que je traduis l'article 1 du texte de la commission des lois. Deuxièmement, la gestion des eaux de ruissellement ne relève pas de l'assainissement.

avec entrain. L'heure est non plus à déplacer les virgules des lois NOTRe ou MAPTAM, mais à restaurer la liberté communale et les intercommunalités dans leur rôle de coopératives de communes.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, la question de l'eau et de l'assainissement revient une nouvelle fois devant notre assemblée. En février 2017, le Sénat avait clairement exprimé sa volonté de conférer au transfert de ces deux compétences à l'échelon intercommunal un caractère optionnel, c'est-à-dire de faire confiance aux territoires, à leur expérience et à leur savoir-faire. Pourquoi ? n'y avait pas de problèmes particuliers s'agissant de la gestion de ces compétences, mais aussi parce que la quasi-totalité des associations d'élus le demandait et ne comprenait pas que cela leur soit refusé. Souvenons-nous que, dès l'origine, les maires ont été surpris par ce texte. Ils n'ont pas été les seuls au demeurant, le volet « eau et assainissement » ayant été rajouté au projet de loi NOTRe, sans même faire l'objet d'une étude d'impact digne de ce nom. À aucun moment, d'ailleurs, les communes n'ont exprimé une telle demande de transfert, car partout, ou presque, des solutions, très souvent intercommunales, pour le bien de toutes les communes. Les maires n'ont pas attendu la loi pour s'organiser et faire face à leurs responsabilités. Ceux des petites communes ont très tôt compris l'intérêt qu'ils avaient à travailler ensemble, dans des configurations et des périmètres appropriés, centrés sur les services à gérer et les projets à construire. Les solutions choisies ont été pensées et édifiées patiemment, pas à pas, en fonction des réalités locales, de la géographie, de la topographie, de la topologie, bref, des particularités et contraintes naturelles de chaque territoire et des attentes et exigences de leurs administrés. Les communes ont ainsi acquis, chemin faisant, une longue pratique de la coopération en matière de services et de réseaux, pratique qu'on veut à présent passer par pertes et profits. L'expérience, hélas, ne vaut plus grand-chose à l'heure où l'expertise est érigée au rang de vertu première. Et Dieu sait ce que nous devons aux experts ... Nous devrions rappeler à certains, mes chers collègues, que si le rôle des parlementaires est multiple, il est moins de penser à la place des autres que de savoir écouter et comprendre. C'est aussi, entre autres missions, l'un des rôles dévolus à la Conférence nationale des territoires. Cependant, si elle devait être animée de la même manière de voir, de la même façon d'être à l'écoute, gageons qu'elle n'obtiendra pas les résultats attendus et qu'elle sera loin, très loin même, de mériter les vertus que d'aucuns lui prêtent. La loi NOTRe a considérablement bouleversé nos territoires, tout particulièrement les territoires ruraux, où la remise en cause des libertés locales est encore plus mal vécue qu'ailleurs. Cette loi a même contribué à changer très fortement la nature de la coopération intercommunale. Elle est désormais vue moins comme un outil au service des communes, librement choisi par elles, que comme une volonté de mettre ces communes au pas dans une course au gigantisme sans limites. Le groupe de travail que vous avez réuni à plusieurs reprises, madame la ministre, a essayé de trouver des solutions acceptables, au mieux des intérêts de tous. En dépit de vos efforts personnels et de ceux des collègues parlementaires qui le constituaient, dont je ne doute pas un instant de la volonté de travailler utilement pour nos territoires, ce groupe n'est pas parvenu à trouver un accord susceptible d'agréer le plus grand nombre. Au moins Au moins aurions-nous dû étendre la minorité de blocage aux communautés d'agglomération, qui, je le souligne, regroupent près de 7 000 communes rurales. S'il va dans le bon sens, cet accord ne va pas assez loin dans le respect des libertés locales. Voilà pourquoi je choisis, pour ma part, de soutenir le texte de la commission des lois, sachant que cette position ne fait pas l'unanimité au sein de mon groupe.

Cela dit, une chose est sûre, nous devons assumer nos responsabilités face à une question importante pour de nombreux territoires, d'où remontent les difficultés de mise en oeuvre d'un texte qui s'impose à eux aujourd'hui. Il importe donc de revenir au fond sans être dogmatique pour prendre en compte la réalité des territoires. Le fond, ce sont d'abord les objectifs du transfert de compétences rationaliser le secteur par rapport à l'usager et au consommateur ; permettre la réalisation d'infrastructures qui répondent aux enjeux de la qualité de l'eau et de la gestion de la ressource

à être un peu pragmatique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas mettre du sens dans le pragmatisme. Pour arriver à une compétence unique et permettre une politique publique de l'eau et de l'assainissement qui ait du sens, cela suppose un long chemin, des études, des diagnostics, des mesures transitoires, des plans d'investissement pour mettre à niveau, une prise en compte des logiques de bassin et des choix de mode de gestion.

Quels sont ces assouplissements incontournables pour nous ? Délai repoussé à 2026, à condition que soit prévu un droit d'opposition au transfert avec le mécanisme de la minorité de blocage extension aux communautés d'agglomération, parce que bon nombre d'entre elles sont aujourd'hui des communautés semi-rurales ; assouplissement du mécanisme de représentation-substitution dans des syndicats élargis ; sécabilité de la compétence « eau-assainissement-SPANC-eaux pluviales » ; enfin, alignement des dispositifs financiers, notamment concernant les agences de bassin, sur ces aménagements à venir. C'est sur cette base que nous avons travaillé sur le texte proposé par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le rapporteur nous propose de revenir à une compétence optionnelle, purement et simplement. Nous ne sommes pas sûrs que cela soit la meilleure manière de servir les territoires que nous représentons et qui fondent notre légitimité. Le plus important pour nous, c'est d'aller dans le sens de l'efficience de la gestion de l'eau, de l'assainissement, en assurant une gouvernance maîtrisée par les acteurs publics Madame la ministre, vous disiez avec le sourire que les petits ruisseaux faisaient les grandes rivières ; j'ose vous dire qu'il arrive que certains se noient dans une flaque d'eau Il semble que le scénario écrit pour cet après-midi risque d'arriver à ce résultat, ce qui est bien dommage pour les territoires que l'on prétend représenter.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement, c'est le terrain, et lui seul, qui enseigne la gouvernance la plus pertinente. La demande des élus, en particulier des élus ruraux, est simple : laisser la liberté aux communes de décider ou non du transfert des compétences « eau » et « assainissement ». Et cette liberté ne doit être ni encadrée, ni limitée, ni transitoire Or le contenu initial de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui ne répondait toujours pas aux préoccupations de nos territoires ruraux. Aussi, je me réjouis que cette proposition de loi ait été profondément remaniée par notre commission des lois, afin qu'elle corresponde au texte déjà adopté à la quasi-unanimité par le Sénat le 23 février 2017, texte qui visait à maintenir les compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes. Cette proposition de loi n'a pas été jugée satisfaisante par la commission des lois du Sénat pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle maintient le caractère obligatoire du transfert des compétences « eau » et « assainissement », et permet seulement de différer son entrée à la condition de réunir au moins 25 % des communes membres d'une intercommunalité représentant au moins 20 % de la population. Ensuite, elle n'englobe pas les communautés d'agglomération, dont certaines ont été créées dans des territoires ruraux. Enfin, la gestion des eaux pluviales et du ruissellement dans les zones urbaines a été incluse dans la compétence « assainissement » des communautés de communes et d'agglomération. La commission des lois a donc confirmé la position adoptée à la quasi-unanimité par le Sénat le 23 février 2017. En premier lieu, elle a voulu pérenniser le caractère optionnel des compétences « eau » et « assainissement » pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, en supprimant le dispositif de minorité de blocage prévu dans le texte de l'Assemblée nationale. En second lieu, elle a souhaité permettre aux communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération de continuer à prendre en charge la gestion des eaux pluviales en cas de transfert de la compétence assainissement » à leur intercommunalité, afin d'apporter une souplesse permettant de mieux prendre en compte les spécificités des situations locales. Je tiens, à cette tribune, saluer le travail accompli par le rapporteur, notre collègue François Bonhomme, qui s'est montré particulièrement attentif aux préoccupations de nos territoires. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants- République et Territoires votera en faveur de cette proposition de loi ainsi modifiée par la commission des lois du Sénat.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte, c'est le festival des hypocrites ! En effet, si on refait l'historique, d'où provient le problème ?

Eh bien, mes chers collègues, cette loi NOTRe a été votée au Sénat par quasiment tout le monde puisque nous n'avons été que 49 sur 348 à voter contre

Mes chers collègues, si l'on veut que le Parlement soit crédible, il ne faut pas

il amortit un tout petit peu les aspects très négatifs de la loi NOTRe, que d'autres ont votée

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution proclamant que le droit à une eau potable et à l'assainissement est un droit fondamental. Dans notre pays, la question de l'accès à l'eau potable est apparue au XIX siècle, en pleine révolution industrielle. Les communes se sont saisies de ces missions, qui constituent l'un des fondements de l'action communale. Il est d'ailleurs opportun de rappeler que l'équipement en réseaux d'eau- tout comme l'électrification -est à l'origine des premières formes de coopération intercommunale. Je pense notamment à la loi du 22 mars 1890 instituant les syndicats intercommunaux à vocation unique. Je rappelle néanmoins que cette coopération se faisait- à l'époque -sur la base du volontariat et sur l'initiative des communes. Au fil du temps, les évolutions institutionnelles, mais aussi la technicité accrue de ces missions, ont abouti à une diversité d'organisation sur l'ensemble de notre territoire où cohabitent plusieurs modes de gestion et où l'on compte un grand nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes. Sans doute trop ! Il en résulte une situation contrastée dans laquelle coexistent un grand nombre de collectivités ou de groupements gestionnaires d'une ou de plusieurs de ces compétences, en totalité ou en partie. La progression des exigences environnementales, la question des rendements ou celle de la qualité de l'eau poussent à une réduction des syndicats ou à une gestion à plus grande échelle, mais posent, en corollaire, la question du coût pour le citoyen. C'est dans ce cadre qu'est intervenue la loi NOTRe prévoyant une réforme radicale, pour ne pas dire brutale, dont cet hémicycle garde en mémoire les intenses débats qu'elle a occasionnés. Je n'y reviens donc pas. Je rappelle néanmoins notre position constante : l'eau a sa propre géographie. Vouloir aligner les communes ou les syndicats d'eau sur les limites des intercommunalités constitue par conséquent une erreur. Très bien ! Cela est d'autant plus vrai dans les territoires de montagne, que je connais bien. Cette loi NOTRe a été adoptée il y a près de trois ans. Elle ne constitue pas un texte immuable et des aménagements ont, depuis lors, été apportés. S'agissant des missions relatives à l'eau et à l'assainissement, la proposition de loi de nos collègues des groupes Les Républicains et Union Centriste, adoptée en février 2017, visait, entre autres, à revenir sur le caractère obligatoire de ces transferts de compétences. Je partage le sentiment exprimé en commission des lois sur le mépris de la majorité à l'Assemblée nationale, qui aurait pu amender ce texte, plutôt que de l'enterrer- nous aurions, en outre, gagné un temps précieux. Nous aurions à redire également sur la forme du présent texte, censé répondre à l'engagement pris par le Premier ministre devant le congrès des maires. Cela étant dit, notre qualité de législateur doit nous conduire à nous interroger sur la meilleure solution pour nos territoires, et plus encore nous, sénateurs, qui assurons la représentation des collectivités. C'est la raison pour laquelle nous avons privilégié une approche pragmatique qui permet des avancées au profit des collectivités concernées, en étant à l'écoute des élus locaux. Que nous disent-ils ? Que les intercommunalités ont été confrontées à des réformes d'ampleur, ces dernières années. Elles se sont vues confier nombre de nouvelles compétences. Elles ont, en outre, vu leur périmètre grandement modifié. Beaucoup nous disent que 2020, c'est trop tôt et qu'elles ne pourront pas procéder à l'harmonisation des modes de gestion dans de bonnes conditions. Ainsi guidés, nous avons proposé plusieurs aménagements au texte adopté par l'Assemblée nationale qui pourraient être de nature à être repris et à faire consensus. Le premier consiste à élargir le dispositif de minorité de blocage aux communautés d'agglomération. une amélioration, concerne la sécabilité de la compétence « assainissement ». Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait que si une communauté de communes avait déjà partiellement transféré une compétence, elle ne pouvait bénéficier du mécanisme de report à l'horizon 2026. Or nous savons que de nombreux EPCI ruraux ont fait le choix de mutualiser l'assainissement non collectif, avec le service public d'assainissement non collectif, le SPANC, tout en maintenant l'assainissement collectif dans les compétences municipales. Cette distinction s'expliquait par le fait que ces deux volets de l'assainissement mobilisent des expertises et englobent des missions distinctes. Cet aspect est d'ailleurs bien expliqué dans le rapport de notre collègue François Bonhomme, que je tiens à remercier de son travail. Enfin, je veux aborder la thématique des eaux de pluie et de ruissellement. Nous en avions déjà débattu dans le cadre de la proposition de loi relative à la GEMAPI.

mixte paritaire lors de la loi GEMAPI me semblait clair. Le Gouvernement devait remettre un rapport sur cette question dans les deux mois suivant la publication de la loi, lequel devait éclairer notre travail législatif. Près de quatre mois après l'adoption de ce texte, le Gouvernement n'a pas tenu cet engagement. Nous aurons l'occasion de nous attarder plus longuement sur ces problématiques lorsque nous aborderons l'examen de l'article 2. Comme ils l'ont fait en commission, les sénateurs du RDSE demeureront fidèles à leur volonté que nous aboutissions, à la fin de la navette parlementaire, au meilleur texte possible pour nos territoires et nos communes. Notre vote sur l'ensemble dépendra donc du sort réservé aux amendements déposés.

pour revenir à une compétence optionnelle, c'est que la compétence « eau », plus encore que la compétence « assainissement », ne répond pas à la seule logique intercommunale. L'eau est liée à une problématique

Pourquoi persistez-vous dans votre vision jacobine ? Pourquoi ne faites-vous pas confiance aux élus locaux ? Le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux intercommunalités est encore un malheureux exemple que, du haut de la capitale, la réalité du terrain est ignorée Du haut de votre Capitole, vous remettez en cause les libertés et la libre administration des collectivités locales ! Le climat s'est détérioré entre les élus et l'État ! Madame la ministre, les élus sont en colère. Vous ne leur donnez pas les bases d'un climat de confiance. En engageant un effort budgétaire bien plus important que l'État ces dernières années, les élus ont très largement démontré qu'ils étaient capables de gérer. capables de gérer. Souhaiter regrouper et rationaliser l'action publique, pourquoi pas ? Mais à marche forcée contre les réalités et les spécificités de nos communes, c'est non Pourquoi persistez-vous à vouloir transférer coûte que coûte ces compétences ? En effet, si la loi NOTRe a prévu que les compétences « eau » et « assainissement » seraient transférées à titre obligatoire aux intercommunalités au 1 janvier 2020, déjà, lors de la discussion de ce texte, les débats avaient montré qu'imposer ce transfert obligatoire relevait d'une vision technocratique et non d'une vision pragmatique de la réalité du terrain. Le Sénat a ainsi proposé de redonner la liberté à nos élus et de décider en fonction des contraintes de leurs territoires. Vous avez préféré renvoyer aux oubliettes cet appel des territoires. Face aux réelles inquiétudes de nombreux élus, le Président de la République s'est engagé, lors du dernier congrès des maires, à revenir sur le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux intercommunalités. Votre gouvernement a présenté un texte afin de modérer ce transfert obligatoire, mais il est clairement en deçà des besoins du terrain et des promesses faites devant des milliers de maires. J'ai participé au groupe de travail que vous avez mis en place afin de faire des propositions pour revenir sur ce transfert. L'espoir est né qu'un équilibré soit trouvé, malgré les difficultés à s'accorder. Et quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que la minorité de blocage avancée comme solution de compromis n'était plus prévue pour les communautés d'agglomération Le Gouvernement est-il, une fois de plus, en train de ne pas respecter sa parole, comme il l'a fait avec l'annonce de l'arrêt de la baisse des dotations, alors que 22 000 communes voient Madame la ministre, permettez-moi de vous rappeler les réalités de notre pays. Il faudrait qu'elle les connaisse ! Véritable échelon de proximité, nos communes sont souvent les mieux placées pour appréhender l'échelle pertinente de mutualisation des services. Plus particulièrement, pour les compétences « eau » et « assainissement », elles sont les mieux à même d'organiser efficacement leur exercice, en fonction notamment des caractéristiques de la ressource. Cela est d'autant plus démontré en milieu rural et en zone de montagne où les contraintes sont plus fortes. Madame la ministre, le rat des champs ne fait pas de bruit pour rien ! S'il invite le rat des villes à venir chez lui, c'est pour qu'il retombe les pieds sur terre et voit comment est le monde au-delà des faubourgs Il apparaît évident, comme le clament nos élus locaux, que le texte que vous nous avez proposé est très insuffisant. Il est préférable, comme le redemande le Sénat aujourd'hui, que l'eau et l'assainissement restent des compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération et qu'aucune date butoir ne soit prévue. En revanche, si vous persistez à ne pas nous écouter, des points essentiels devront être ajoutés à votre texte. Tout d'abord, les communautés d'agglomération doivent pouvoir aussi déroger au transfert des compétences « eau » et « assainissement », avec le mécanisme de la minorité de blocage. En effet, d'une part, à ce stade, 48 % des communautés d'agglomération n'ont pas la compétence « eau D'autre part, pour les territoires ruraux, la taille de certaines communautés d'agglomération est comparable à celle des communautés de communes. Votre proposition de loi crée ainsi une rupture d'égalité entre les communes selon la nature de l'intercommunalité à laquelle elles appartiennent.

? Enfin, il est essentiel de scinder la gestion des eaux pluviales de la compétence « assainissement ». Son transfert est particulièrement complexe et peut être rattaché à plusieurs compétences, à la voirie, par exemple. Pour Pour conclure mon propos, je souhaite vous faire part de mon désaccord avec les arguments de ceux qui soutiennent obstinément l'obligation du transfert de ces compétences. Avancer que la qualité de l'eau serait améliorée est une vue de l'esprit ! Si cela consiste à tout traiter, cela ne sert à rien Prétendre que tous les investissements nécessaires seraient faits est une véritable supercherie ou alors relève du miracle, dans un contexte de baisse des subventions ! Quant à l'harmonisation administrative des tarifs, elle conduirait à une forte augmentation du prix de l'eau dans les territoires ruraux, où l'on peut craindre que tout cela ne finisse dans les mains de grands groupes qui imposeront des tarifs que les élus ne pourront plus maîtriser. Alors, madame la ministre, écoutez et entendez nos élus locaux, qui aujourd'hui n'ont plus confiance et qui attendent de vous tout simplement un peu de bon sens

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, chers collègues, l'eau, nous le savons tous, est une ressource naturelle vulnérable et extrêmement fragilisée par des pollutions de toutes origines. Et les débats sur l'eau doivent toujours être replacés dans ce contexte et dans la perspective des générations futures. Il est donc légitime que la question de sa gestion soit posée. Quelle est la situation aujourd'hui ? Le droit actuel prévoit le transfert obligatoire aux intercommunalités, au 1 janvier 2020, des compétences relatives à l'eau potable, aux eaux usées La réalité, c'est aussi des modes de gestion sur le terrain très disparates, avec des problématiques complètement différentes entre le secteur rural et le secteur urbain. Trois hypothèses s'offrent à nous. on reste dans le droit actuel de la loi NOTRe, voulue par le gouvernement précédent. Nous le savons, il serait alors impossible, pour bon nombre d'intercommunalités, de réussir ce transfert dans de bonnes conditions, au 1 janvier 2020. Deuxième hypothèse, on revient au texte voté par le Sénat en février 2017 qui faisait le choix de la compétence optionnelle- ce que propose finalement la commission. Je comprends cette position, qui est en cohérence avec le vote de l'an passé

et nous savons tous qu'il n'a pas plus de chance d'aboutir cette année. Nous sommes donc dans une impasse. Pour ma part, je ne pense pas qu'il soit opportun de nous arc-bouter sur un texte qui nous conduirait dans une voie sans issue.

la procédure de la minorité de blocage, et ce jusqu'en 2026. Telle est la solution qui a été adoptée par la grande majorité des groupes à l'Assemblée nationale. Avec plusieurs collègues du groupe Union Centriste, nous adhérons à cette solution de compromis, qui laisse aux collectivités le temps de se préparer sereinement. nous vous demandons, de votre côté, madame la ministre, d'accepter des améliorations au texte de l'Assemblée nationale sur deux points importants. Première amélioration, la sécabilité de la compétence « eaux pluviales » sans limitation dans le temps. La gestion des eaux de ruissellement dans le secteur rural doit demeurer une compétence communale. Le bon sens du terrain l'exige. Priver les communes de cette maîtrise compliquerait inutilement la gestion quotidienne des eaux de ruissellement et pénaliserait les projets d'aménagement de bourgs ou de villages. Seconde amélioration importante, la possibilité de dissocier jusqu'en 2026 les compétences « assainissement collectif » et « assainissement autonome ». Pourquoi ? Parce que le zonage en assainissement autonome est très présent dans le milieu rural. Et cette compétence -a souvent été transférée aux communautés de communes sans que, pour autant, la compétence de l'assainissement collectif ait été transférée. Or la loi NOTRe prévoit que la compétence « assainissement » est globale sans pouvoir dissocier l'assainissement collectif de l'assainissement autonome. Nous vous demandons, madame la ministre, de veiller particulièrement à ce point, qui pourrait conduire- ce serait un comble ! -les intercommunalités rurales détenant la compétence du SPANC à se voir imposer la compétence de l'assainissement collectif dès le 1 janvier 2020, alors même que le report à 2026 aurait été adopté par le Parlement. Je vous demande vraiment d'éviter cette situation absurde ! Enfin, je tiens à vous remercier, madame la ministre. En effet, nous étions face à un blocage et vous avez joué un rôle important dans le déblocage de ce dossier. Dans un contexte que je sais compliqué, vous apportez une réponse concrète à une situation qui semblait inextricable.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans cet hémicycle, nous en appelons souvent à la nécessité de simplifier notre législation, de la rendre plus facilement compréhensible et applicable pour les élus locaux qui la mettent en oeuvre et en mesurent les effets. Des effets qui ne sont pas toujours positifs ou conformes aux intentions initiales du législateur. Parce que les élus le demandaient, le Gouvernement a donc engagé un travail de simplification de la loi NOTRe pour son volet « eau et assainissement C'est une bonne initiative ! Avec mon collègue Jean-Yves Roux, que j'associe pleinement à cette expression, le groupe socialiste et républicain a fait des propositions constructives au sein du groupe de travail. À l'écoute de nos territoires et de leurs élus, nous avons fait valoir les principes et positions suivants : d'abord, desserrer la contrainte de la loi en abaissant le seuil minimal du nombre d'EPCI regroupés en syndicat de trois Cette disposition évitera de supprimer des structures qui ont parfois fait la démonstration de leur efficacité et qu'il est souhaitable de préserver dans leur organisation actuelle. Ensuite, laisser aux élus locaux le temps de procéder à des études technico-économiques sur un laps de temps pluriannuel, selon des scénarii multiples intégrant les dépenses et recettes actualisées des différents postes de coûts. Ces études permettent d'apprécier dans le temps le niveau et les évolutions du prix et de la qualité du service rendu et de choisir le scénario optimal pour l'usager. pour permettre aux élus de mener à bien ces études, nous proposons de repousser l'échéance butoir pour le transfert de compétences à 2026, en gardant jusque-là le caractère optionnel de ces compétences. Nous sommes donc favorables à ce que la minorité de blocage du transfert puisse être exercée, l'intérêt que nous y voyons étant de permettre aux élus d'arriver à construire progressivement un consensus rationnellement étayé avant l'échéance de 2026. Pour coller le plus possible à la réalité du terrain et prendre en compte les différences de problématique entre eau, assainissement, ruissellement et eaux pluviales, nous pensons aussi utile que la sécabilité des compétences soit effective.

Nous souhaitons en outre que les démarches déjà engagées sur les territoires ne soient pas remises en question par les décisions que nous allons prendre en légiférant. Je veux aussi rappeler que la loi actuelle, sur un périmètre de syndicat donné,

L'uniformisation du mode de gestion et l'égalité tarifaire peuvent ainsi être évaluées en tant que stratégie planifiée dans le temps si les élus le souhaitent pour et avec les usagers. Un autre point mérite attention parce qu'il touche à l'engagement citoyen comment préserver, dans le cadre adapté que nous allons définir, la participation actuelle de conseillers municipaux ou de délégués des communes au sein de syndicats ou de régies existants amenés à disparaître, alors que ces personnes ne sont pas conseillers communautaires ? Le service de l'intérêt général par ces citoyens actifs et dévoués s'en trouverait affaibli. Il faut l'éviter, et cela mérite que nous en discutions. Pour terminer, Jean-Yves Roux et moi-même voulons saluer l'intention initiale qui a présidé aux travaux du groupe piloté par Mme la ministre Jacqueline Gourault. La suite nous a pour le moins surpris, avec une proposition de loi du groupe majoritaire de l'Assemblée nationale plutôt qu'un projet de loi gouvernemental et un débat législatif qui commence à l'Assemblée nationale pour un texte relevant de l'organisation des collectivités locales.

que nous entreprenions de telles démarches sur d'autres sujets ; je pense en particulier à l'urbanisme. Mon dernier mot sera en forme de voeux, pour aujourd'hui et pour demain : ne refaisons pas, sur le sujet de l'eau, le débat de la loi NOTRe ! Adaptons pragmatiquement ce qu'elle est aujourd'hui, en ayant en tête de donner plus de liberté aux élus locaux, dans l'intérêt premier des populations et des territoires ! La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la loi NOTRe a suscité de nombreux débats. Plus de deux ans après son adoption, elle soulève encore des questions et des doutes. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise- je l'espère -à conclure ces débats qui n'ont que trop duré.

de réaliser des économies d'échelle, d'augmenter les capacités d'investissement et ainsi d'harmoniser les prix. Certes, ces avantages ne sont pas négligeables, mais ils n'ont pas suffi à rassurer les acteurs concernés. En effet, le débat s'est crispé sur l'aspect contraint du transfert de compétences qui a été très mal perçu. Nous touchons ici à l'essence même du principe de la libre administration des communes, auquel nous sommes tous dans cette enceinte profondément attachés. Imposer une obligation aux collectivités apparaît dès lors contraire à ce principe. faut par conséquent laisser aux élus locaux une certaine liberté, parce qu'ils sont légitimes et, surtout, parce qu'ils sont les seuls à avoir une connaissance suffisante du terrain pour déterminer la meilleure option à retenir. Pour répondre à ces inquiétudes locales, certains sénateurs ont souhaité maintenir les compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération ; ils ont, à cette fin, déposé une proposition de loi en janvier 2017. Une fois adoptée par le Sénat à la quasi-unanimité, elle avait été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en octobre 2017. Le texte a toutefois fait l'objet d'une motion de renvoi en commission ; je le regrette. Madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous allons discuter a été profondément remaniée par notre commission des lois, afin qu'elle corresponde au texte déjà adopté par le Sénat en 2017.

et pourquoi nous lui préférions celui qui avait été adopté à la quasi-unanimité dans cet hémicycle. J'en profite pour le féliciter pour son excellent travail. Au-delà des aspects techniques, l'obstination du Gouvernement à vouloir conserver l'article 64 de la loi NOTRe soulève une question pourquoi cette obsession à vouloir vider de leurs compétences les communes, cellules de base d'une République dite décentralisée ? Cet échelon de proximité est un atout pour les enjeux liés à la ruralité. Or la loi NOTRe, en redistribuant ces compétences de manière dogmatique, aura eu des conséquences très négatives pour les communes rurales. Les intercommunalités de taille déraisonnable sont des schémas artificiels qui ne sauraient se calquer par magie sur les réalités si différentes de nos territoires. L'eau et l'assainissement, au même titre que l'urbanisme, figurent parmi les compétences essentielles de nos villes et de nos villages. Après leur disparition, que restera-t-il aux communes pour organiser leur destin commun ? Rien, mis à part la médiation des conflits de voisinage, la présidence du repas communal des personnes âgées et la gestion du cimetière ! Avec le texte adopté par l'Assemblée nationale, nous dépassons cette fois toutes les lignes rouges.

se sont tenus lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, j'ai découvert avec intérêt que bien des députés de la majorité, qui se flattent d'être vierges de tout antécédent électoral et de l'exercice d'un mandat local, claironnent que le transfert de ces compétences aux EPCI créera des économies d'échelle. Ils sont coupés des réalités ! Or chaque maire qui a travaillé sur l'intégration intercommunale connaît les problèmes d'apparition de doublons dans les effectifs, et sait aussi que l'intercommunalité à marche forcée rime avec une hausse des coûts globaux de fonctionnement que l'État vient ensuite montrer du doigt. Tout à fait ! Si le transfert de compétences est source d'économies dans certains cas, c'est tant mieux, et faisons-le ! Mais c'est, hélas, l'effet inverse qui se produira dans beaucoup d'autres situations. Tandis que la commune assurait la distribution de l'eau avec des moyens humains limités et peu coûteux, l'organisation à l'échelle de l'intercommunalité nécessitera un affermage, qui sera vraisemblablement concédé à de grandes sociétés privées, ce qui fera mécaniquement augmenter les coûts pour les utilisateurs. Ce sera notamment le cas dans les territoires de relief et, particulièrement, dans la montagne ardéchoise, que je connais bien et dont je pourrais vous parler longuement. La communauté de communes de la Montagne

Depuis toujours, chaque commune de ce territoire a organisé sa propre distribution d'eau, et ce à un prix modeste, malgré les difficultés liées au relief. Madame la ministre, vous connaissez aussi bien que nous les élus locaux lorsqu'une mutualisation des moyens était pertinente, ils n'ont pas attendu le vote d'une loi pour s'organiser à un échelon efficient et monter des syndicats. Laisser la compétence aux communes qui le désirent est indispensable, mais à condition qu'elles en aient les moyens. C'est pourquoi j'ai signé et je soutiens l'amendement n° 23 rectifié, déposé par ma collègue Patricia Morhet-Richaud, qui vise à préciser que les communes restent éligibles aux diverses aides publiques. Sinon, sans moyens financiers, le transfert deviendra obligatoire. C'est d'ailleurs aussi l'occasion, peut-être, de s'interroger sur la raison d'être des agences de bassin, qui ne soutiennent plus les communes, en particulier, les plus petites Je terminerai mon propos en rappelant un point essentiel : 21 % des communes rurales sont intégrées à des communautés d'agglomération ou à une métropole. Elles ne sont même pas mentionnées dans ce texte, alors qu'avec elles 5 millions de nos concitoyens sont de fait privés de la capacité de décider de leur propre sort ! La parole

Ce document est paru il y a quelques jours ; il est en cours de transmission au Parlement.

! Selon lui, la taxe GEMAPI pouvait répondre, en partie seulement, au problème du ruissellement dans les zones rurales.

la compétence « assainissement » entre le SPANC et le collectif. En revanche, j'ai bien entendu,

le processus législatif qui a été suivi jusqu'à présent. Madame la ministre, je dois dire que, sur toutes les travées de cet hémicycle, les membres du Sénat ont été étonnés, surpris et, pour certains, même choqués

d'usage pour les textes concernant les collectivités territoriales. Qui plus est, cette proposition de loi ne fait qu'une partie du chemin nécessaire pour apporter une réponse concrète à nos collectivités. Tout cela

pour cette procédure et pour le mépris dont le Sénat a pu faire l'objet dans l'étude de cette question délicate, mais aussi mon souhait que le Sénat confirme son vote de l'année dernière.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je crois au temps long et à l'inscription de nos décisions dans ce temps long. Or, en matière d'approvisionnement en eau et de traitement de cette la loi NOTRe, comme la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, tout particulièrement, son article 1 dans sa version initiale, ainsi que certains amendements déposés au Sénat à cet article sont en rupture avec notre histoire, car ils tournent le dos aux libertés communales. L'histoire de l'approvisionnement en eau est en effet celle de constructions qui, quoiqu'extrêmement diverses, ont globalement donné la part belle à l'échelon communal. Communes et syndicats ont su, au fil du temps, s'adapter à la géographie locale et élaborer des systèmes ingénieux et performants de distribution et de traitement de l'eau. Dans notre vieux pays jacobin, c'est presque un contre-exemple qui s'est imposé, loin des schémas d'uniformisation. Dans les zones de montagne comme dans les territoires les plus éloignés, la liberté qui a été donnée aux élus a permis une couverture exceptionnelle de notre pays par des réseaux efficients. Cela ne fut possible que par l'engagement bénévole de nombreux élus : ils étaient persuadés de concrétiser là leur volonté de s'engager pour un service public de qualité et au meilleur prix pour tous les usagers, jusqu'à ceux qui étaient les plus éloignés des grands centres urbains. revanche, la rationalisation qui nous est proposée aujourd'hui n'est que le faux nez de la centralisation. Certes, aucun système ne peut rester figé. Tout le monde en convient, et l'importance des investissements peut militer pour la recherche d'une taille critique. Mais les collectivités n'ont pas attendu la loi NOTRe pour aller dans ce sens, celui d'une gestion efficace et responsable ! Lorsque cela était souhaitable, les EPCI se sont organisés pour optimiser la gestion de l'eau. eux exercent déjà cette compétence. C'est bien la preuve que les élus locaux n'ont pas de position dogmatique et savent choisir la meilleure option. Madame la ministre, mes chers collègues, il y a dans le domaine de l'eau autant d'histoires, autant d'engagements bénévoles et autant de constructions que de territoires.

l'exercice de la compétence « eau et assainissement », que nous abordons à travers cet article 1, est un sujet majeur. Il s'agit d'un service public essentiel et vital pour nos concitoyens. Au vu de notre histoire et de la diversité des territoires, la seule réponse que nous pouvons apporter est celle de la confiance dans les élus locaux. Ils ont su, au fil des années, se regrouper entre communes pour mutualiser cette compétence en fonction de diverses contraintes géographiques locales, en conservant toujours le bon sens qui les anime. Grâce à cela, aujourd'hui, 96 % des Français ont accès à l'eau potable, et ce pour un prix inférieur à la moyenne européenne. C'est bien la preuve que les communes sont capables de juger par elles-mêmes s'il est pertinent ou non de transférer cette compétence à l'intercommunalité. Je regrette vivement que la proposition de loi issue des travaux de l'Assemblée nationale, en prolongeant l'esprit de la loi NOTRe, rompe avec cette confiance historique, en particulier à travers son article 1. Alors que des assises de l'eau sont annoncées pour cette année, il aurait été cohérent d'aller dans le sens d'une plus grande liberté pour les communes et de continuer à faire confiance à leurs savoir-faire. Malheureusement, le texte de l'Assemblée nationale nous propose le contraire, en introduisant la date butoir de 2026, et ce sans qu'aient été consultés les sénateurs du groupe de travail compétent, alors qu'un compromis avait pourtant été trouvé. Pour ma part, je considère que ne pas donner écho à ce texte est une grave erreur. Et puis certains esprits tourmentés pourraient y voir une sorte de mépris à l'égard des élus. Enfin, je veux rappeler un point important. L'extension du périmètre de la compétence implique aussi le passage d'une gestion de proximité à une gestion par des organismes extérieurs.,

pour conserver une politique de l'eau adaptée aux contraintes des territoires, et ce à des coûts constants pour nos concitoyens. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le texte dont nous débattons aujourd'hui soulève la question de notre conception de l'efficience de l'action publique. L'eau et l'assainissement ne sont que des sujets techniques et devraient donc être examinés avec pragmatisme et souci d'efficacité. Or que constatons-nous ?

allait jusqu'à nous laisser croire que la loi pourrait commander aux éléments naturels en rattachant leur gestion à un périmètre administratif ! Ma deuxième remarque est tout à la fois un constat et un regret, ceux d'un dialogue très difficile entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur un sujet technique qui concerne nos collectivités, dont le Sénat est le représentant. Le rejet par l'Assemblée nationale de la proposition de loi sénatoriale empreinte de pragmatisme et d'efficacité, adoptée ici à l'unanimité, résonne comme l'affirmation d'une vision technocratique et d'une absence de confiance dans les élus locaux et leur sens des responsabilités. Ce sujet a ainsi été totalement pollué, ce qui est un comble quand on parle de qualité de l'eau Je salue, madame la ministre, avec beaucoup de respect et de sincérité, votre engagement sur ce sujet ... À juste titre ! ... et votre volonté de sortir d'une longue errance née de la loi NOTRe. Vous avez réussi à construire une issue à une impasse née du rejet de la position du Sénat qui consistait à permettre plutôt qu'à imposer. Toutefois, pardonnez-moi, cette issue ressemble à une sorte de liberté conditionnelle, du fait de la minorité de blocage. En cohérence avec l'attente des élus de mon territoire, je vous confesse que j'aurais préféré une vraie liberté de faire, selon que l'efficacité l'exige ou non. La parole

pour les intercommunalités qui exercent de façon partielle la compétence « eau et assainissement » sur leur territoire, de sorte que les autres communes puissent continuer à exercer une compétence individuelle. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini,

La proposition de loi donne la possibilité aux communes membres de communautés de communes qui n'auraient pas déjà transféré leurs compétences « eau » et « assainissement » de s'opposer au transfert de ces compétences avant le 1 juillet 2019,

la problématique est, non pas la date du transfert de compétences, mais bien son caractère obligatoire, fût-il décalé dans le temps. On ne peut pas aborder la gestion de l'eau et de l'assainissement de manière dogmatique et systématique, parce que ces problématiques s'ancrent nécessairement dans la diversité de nos territoires. Si je ne siégeais pas à vos côtés à cette date, mes chers collègues, je partage néanmoins totalement la position adoptée à l'unanimité par le Sénat le 23 février 2017. Loin des dogmes et des conjectures, je veux répéter dans cet hémicycle qu'il y a une vie territoriale, des compétences et du professionnalisme au-delà des espaces métropolitains. Cela se vérifie particulièrement pour les questions d'eau et d'assainissement, même si ces deux questions pourraient être différenciées. Chaque jour, dans nos communes, des élus travaillent bénévolement et avec un haut niveau d'exigence. Chacun de nous aurait des histoires à raconter pour témoigner de ces élus bénévoles, qui se mettent au service de tous et qui, de surcroît, permettent de limiter le prix du mètre cube d'eau. Je ne suis pas opposé aux regroupements de communes qui permettent de mieux organiser et de mutualiser nos moyens ; je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai été président de ma communauté de communes et que je l'ai fait fusionner avec la communauté de communes voisine. Bien entendu, il existe localement des difficultés quant à la gestion de l'eau et de l'assainissement. Le transfert de compétence peut apporter une solution. Néanmoins, il existe de nombreux territoires où cette gestion se déroule dans les meilleures conditions et offre un service de qualité à nos concitoyens. Il serait dommageable de casser ces modèles de réussite parce que l'on souhaite calquer et uniformiser un modèle semblable partout. Ne nous trompons pas : la très grande majorité des élus locaux savent organiser ces questions en fonction des contraintes et des atouts

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j'ai voté la proposition de loi du mois de février 2017 et je suis favorable au retour au caractère optionnel de ces compétences- j'avais d'ailleurs déposé un amendement en ce sens en commission. La loi doit laisser les élus communaux décider quelle est la meilleure solution pour la gestion de l'eau potable et de l'assainissement sur leur commune. Nous savons que, pour des raisons topographiques ou historiques, les situations locales sont trop différentes pour qu'un modèle puisse être appliqué partout avec la même efficacité, et ce dans l'intérêt des citoyens. Que je sache, le fait que ces compétences soient optionnelles n'empêche pas- et n'a d'ailleurs pas empêché -les EPCI et les communes qui le souhaitent de réaliser ce transfert. Madame la ministre, beaucoup d'élus que je rencontre voient dans une méconnaissance peut-être -de ce qu'ils sont parvenus à mettre en oeuvre, souvent au prix de nombreuses heures de disponibilité et de travail bénévole, pour que les services de l'eau et de l'assainissement soient rendus de la manière la plus efficace et la moins coûteuse. Pour nombre d'élus ruraux, l'obligation de transférer ces compétences, que ce soit en 2020 ou, plus tard, en 2026, apparaît comme le dernier assaut contre les fondements de la commune. Un maire m'a dit tout récemment : « Vous savez, si je perds la gestion de l'eau, je ne connaîtrai plus les habitants de ma commune, car c'est le dernier lien social qui nous reste.

et devront rapidement harmoniser les modes de gestion pour atteindre une certaine équité sur leur territoire. À ces échelles, la maîtrise de la ressource en eau et des coûts de gestion est moins bien assurée qu'à l'échelon d'une commune ou d'un syndicat de communes à taille humaine. Cela paraît d'autant plus vrai lorsqu'on connaît le fonctionnement des grands groupes en matière tant de recherche et de réparation des fuites que de rentabilité, laquelle nécessite par exemple des hausses de tarif pour compenser des consommations rendues plus faibles par les comportements plus économes des citoyens. Chaque fois que j'interroge des maires de la Drôme sur le réseau d'eau et d'assainissement, je suis surprise du niveau de modernisation. Contrairement à ce qui est généralement avancé, les investissements ont été réalisés sans qu'il soit besoin de transférer la compétence. C'est pourquoi je suis définitivement favorable à ce que les compétences « eau » et « assainissement » soient optionnelles pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération.

Élus ruraux, nous sommes attachés au fait de pouvoir continuer à mener des politiques locales de préservation de la ressource en eau et du cycle de l'eau avec des investissements en rapport. Force est de constater que, dans certains territoires, compte tenu des difficultés géographiques, topographiques, climatiques supplémentaires, certains investissements indispensables ne sont pas envisageables. Certains investissements nouveaux- je pense au recours au traitement de données informatisées -ne pourront pas non plus être assurés sur l'ensemble de nos communes. Mes chers collègues, l'essentiel aussi, en termes de méthode, est à mon sens de préserver la décision des exécutifs communaux. La minorité de blocage temporaire qui a été proposée à l'issue du groupe de travail est intéressante, d'autant qu'elle se calque sur une solution qui a déjà été arrêtée ici même pour le PLUI par le biais d'un amendement de mon groupe. Pour le PLUI, la minorité ne comportait pas de date-butoir, sinon le renouvellement des exécutifs. Je crois que nous aurions pu faire de même, sans grand dommage sur les objectifs à atteindre et tout en préservant la liberté des communes. Nous avons, aujourd'hui plus encore, le devoir de simplifier au maximum toute possibilité dérogatoire que nous pourrions examiner, d'autant examiner, d'autant plus que les communes ont tout fait pour assurer ce transfert dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possible. Nous pouvions difficilement lancer le signal que leurs efforts ont été vains. Pour autant, je tiens à demander au Gouvernement de faire preuve de la plus grande équité pour aider les communes qui le souhaitent à effectuer ces transferts de compétences. En effet, nos communes rurales ont plus que jamais besoin d'une ingénierie pour assurer ces transitions. Madame la ministre, l'intercommunalité choisie nécessite que l'exécutif propose des appels d'offres de grande ampleur, des appels d'offres ciblés, par exemple aux territoires de montagne, très en retard sur l'intercommunalisation. C'est à cette condition aussi que l'équité des territoires pourra être assurée et que le véritable objectif- la préservation efficace de la ressource en eau -pourra être atteint. Je profite également de ce débat pour poser les termes d'une possible péréquation entre les territoires qui doivent faire face à des charges d'entretien de l'assainissement de la gestion des eaux pluviales très différentes. Le volet financement est en effet absent de cette proposition de loi. La parole est à Mme Cécile Cukierman,

eux qui connaissent les contraintes des territoires. À chacun sa solution locale, au plus près des besoins, mais aussi des contraintes et des possibles. On parle sans cesse de simplifier les normes. Alors, simplifions

on a continué à transférer sans discernement ni souplesse de plus en plus de compétences et de pouvoirs des communes vers les intercommunalités. Pour quel résultat ? Une gestion du bloc communal plus coûteuse que par le passé, sans amélioration significative du service rendu.

! Ce que nous contestons, c'est non pas le transfert des compétences, mais son caractère souvent obligatoire. Madame la ministre, dans ce contexte dont vous n'êtes pas totalement responsable, les assouplissements que vous nous proposez sont méritoires, mais nous paraissent insuffisants.

nous voulons le meilleur pour nos collectivités et nos communes, nous allons provoquer le pire, à moins que cela ne relève d'un calcul peut-être plus politique de la favorable à la recherche d'un compromis. C'est la raison pour laquelle, de manière pragmatique, je ne pourrai pas soutenir le texte de la commission. Un coup d'un côté, un coup de l'autre ! La parole est à M. Jean-Pierre Sueur,

« de force » par les préfets. C'est une réalité ! Nous en reparlerons un autre jour. Je tiens à rappeler comment les choses se sont passées. Lors de la commission mixte paritaire sur la loi NOTRe à laquelle je participais, les députés avaient prévu

La loi NOTRe proposait de transférer les compétences susvisées en 2020. Votre proposition, madame la ministre, constitue un progrès non négligeable et nous vous remercions de cette prolongation possible jusqu'en 2026.

nous serions coupables d'être cohérents avec nous-mêmes, avec un texte que nous avons adopté ici même voilà un peu plus d'un an ? Ce serait une victoire à la Pyrrhus, car

dans les meilleures conditions possible le texte sur la GEMAPI, c'était de disposer du rapport qui devait permettre d'introduire des dispositions dans ce texte. Encore

il s'agit d'amendements de principe destinés à dénoncer la nature un peu tordue de certaines règles qui régissent les relations entre les communes et les intercommunalités. L'amendement n° 31 vise à remplacer la minorité de blocage pouvant s'opposer au transfert de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement » par une majorité d'adhésion. La minorité de blocage un mauvais climat, un climat de défiance, au sein d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération. Il est donc préférable d'avoir une adhésion. C'est pourquoi, si une ou plusieurs communes s'opposent, par une délibération prise en conseil municipal, au transfert de l'une ou de plusieurs de ces compétences avant le 1 juillet 2019, il est prévu que les autres communes de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération disposeront de trois mois pour délibérer en faveur de ce transfert ces derniers n'entrant en vigueur que si une majorité de communes représentant au moins 75 % d'entre elles et 80 % de la population délibèrent en ce sens. C'est en quelque sorte l'inversion de la charge de la preuve.

Sans remettre en cause la date butoir de 2026 et en intégrant les communautés d'agglomération au dispositif, il s'agit de prévoir la possibilité pour les communautés de communes ou les communautés d'agglomération n'ayant pas transféré les compétences « et « assainissement », que celui-ci soit collectif ou non collectif, de délibérer entre le 1 janvier 2020 et le 1 janvier 2021 pour organiser ce transfert obligatoire. Les communes membres peuvent s'y opposer, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'alinéa 1, et ce afin d'éviter de plonger les intercommunalités n'ayant pas transféré les compétences « eau » et « assainissement » dans une situation d'instabilité entre 2020 et 2026. Tout en tenant compte du renouvellement municipal et communautaire devant intervenir au mois de mars 2020, nous proposons de définir un créneau d'une année pendant lequel l'intercommunalité peut délibérer pour organiser le transfert obligatoire de ses compétences. Il s'agit d'ouvrir une fenêtre aux intercommunalités voulant se saisir de la compétence, tout en prévoyant une possibilité de blocage pour les communes. Si une telle délibération n'était pas intervenue avant le 1 janvier 2021 ou s'était heurtée à la minorité de blocage dans les conditions prévues à l'alinéa 1, les compétences demeureraient exercées par les communes jusqu'au transfert obligatoire à l'intercommunalité, prévu au 1 janvier 2026. Il s'agit donc de donner pleinement corps à l'annonce faite par le Premier ministre lors du congrès des maires de France.

-de s'opposer au transfert des compétences « eau » et « assainissement », à condition de réunir une minorité de blocage, comprenant 25 % des communes représentant 20 % de la population. En outre, il est précisé que le droit d'opposition est accordé à toutes les communautés de communes, y compris celles qui n'exercent que partiellement la compétence « assainissement ». La question de la sécabilité de la

alors que nombre d'entre elles, comme l'a rappelé notre collègue Mathieu Darnaud, ont une forte dimension rurale, ce qui les apparente plus à des communautés de communes rurales qu'à de véritables communautés d'agglomération.

En outre, vous souhaitez restreindre les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1 de la proposition de loi en limitant la possibilité pour l'EPCI à fiscalité propre de se prononcer sur le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » à une période allant de janvier 2020 au 1 janvier 2021.

explication de vote.

Le scrutin est ouvert.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

« assainissement » de demeurer éligibles aux aides des divers organismes, dont les agences de l'eau, dans le cadre des travaux ou investissements à venir sur leur

la possibilité de demeurer éligibles à l'intégralité des aides des divers organismes, notamment les agences de l'eau, pour les travaux et les investissements futurs. Cette disposition s'inscrit dans l'esprit de l'article 84 de la loi Montagne du 28 décembre 2016 Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence.

Si je l'ai déposé, c'est que je sais combien les élus des communes de montagne sont attachés à la compétence « eau ». Ceux-ci ont installé, par exemple dans mon département et ses vallées pyrénéennes, des systèmes particulièrement adaptés à la montagne et veulent conserver cette compétence.

et validés en conseil d'administration après avis conforme du comité de bassin. Bien sûr, le maintien de l'exercice communal des compétences « eau » et « assainissement » ne remet pas en cause la possibilité la possibilité de percevoir des subventions des agences de l'eau. Je précise que les discussions relatives aux programmes d'intervention relèvent du niveau local et de la disposition locale.

d'une loi qui rassure, en l'espèce, d'une loi qui réaffirme que la règle ne subordonnera pas, demain, à la remontée de compétences le bénéfice des subventions ou aides publiques, quelles qu'elles soient et quelle que soit leur origine,

pour éviter que, demain, les agences de l'eau puissent mettre en place des critères qui conduiraient à empêcher les communes d'accéder à un certain nombre d'aides auxquelles auraient droit les intercommunalités. La mise en oeuvre du dispositif tel

Il convient néanmoins de savoir ce qui est exactement visé. Soit l'on parle d'une régie qui exploite un SPIC ; soit l'on parle d'un service commun d'une collectivité qui exploite, toujours en régie, un SPIC. Dans ce second cas, rien n'interdit à une collectivité, pour des raisons de mutualisation de ressources, de recourir à un service unique pour gérer un SPIC, sous réserve néanmoins que chaque SPIC individualise, sous la forme d'un budget annexe, l'exploitation de chacun des services publics concernés. Cela nécessite toutefois une comptabilité très fine, afin d'analyser les charges relevant de chaque service ainsi que le décompte des équivalents temps plein pour l'exploitation de chacun d'entre eux. L'exploitation d'un SPIC sous la forme d'un budget annexe représente un principe essentiel des finances publiques locales, puisqu'il permet justement d'individualiser les charges et ressources afférentes à ce SPIC.

En revanche, un service unique d'une collectivité peut exploiter, en régie, plusieurs SPIC, dès lors que chacun d'entre eux fait l'objet d'un budget annexe individualisé. Le droit en vigueur ne l'interdit pas, cela relève tout simplement du principe de libre administration des collectivités locales.

laisser le choix, que d'avoir la possibilité de cumuler les deux régies en une seule.

Monsieur le président, mes chers collègues, 20 rectifié vise à sécuriser les régies existantes ou en cours de création exploitant plusieurs services publics à caractère industriel et commercial, administratif, SPA, relatifs aux compétences de distribution d'eau potable et d'assainissement. De nombreuses régies exploitant plusieurs SPIC ou SPA ont été créées par les collectivités locales depuis des décennies, pour le plus grand bénéfice des usagers. Toutefois, depuis quelques années, il semble que prévaut une nouvelle interprétation du cadre légal par l'administration, notamment de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales imposant la création d'une régie pour l'exploitation directe de chaque service public. Cette séparation en deux entités distinctes implique, de fait, de dédoubler un certain nombre de procédures, d'outils, de personnels, induisant des coûts supplémentaires, qui se répercutent sur l'usager, et nuisant à la lisibilité du service public. Aujourd'hui, plusieurs centaines de communes et d'EPCI relèvent d'une régie commune d'eau et d'assainissement. Si leurs régies respectives devaient se scinder en deux, alors le tarif de l'eau ne manquerait pas d'augmenter sur les territoires concernés. Rendre le service public plus efficace et lisible pour les abonnés,

notamment pour la gestion du personnel mutualisé, ces régies communes font sens sur nos territoires. Nous défendrons donc également ces deux amendements et les voterons. Je mets aux

l'établissement d'un budget annexe pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe. Cette disposition a pour objet de permettre la prise en compte de la taille des communes, afin de dispenser les plus petites d'entre elles de l'obligation de suivre, en budget annexe, les activités d'eau et d'assainissement si elles présentent un état sommaire des montants des recettes et des dépenses affectées à ces services. Or l'amendement qui est ici proposé vise à exonérer de l'obligation de suivre, sous la forme d'un budget annexe, les services de distribution d'eau potable et d'assainissement, qui sont des services publics industriels et commerciaux, et à ce titre soumis à un principe, que chacun connaît, d'équilibre budgétaire, avec pour conséquence l'individualisation des dépenses et des recettes dans un budget spécial annexé au budget de la commune ou du groupement de communes.

territoriales, et hors cas spécifiques, il est interdit aux communes de prendre en charge, dans leur budget, des dépenses au titre des SPIC. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement, dont à l'encontre des principes d'équilibre budgétaire et d'individualisation des opérations sous la forme des budgets annexes qui régissent les SPIC, et dont la dispense ne doit concerner que des communes de petite taille, inférieure à 500 habitants. Je vous remercie,

Avant la loi NOTRe, le législateur avait autorisé les communes de moins de 3 000 habitants, mais aussi les EPCI dont aucune commune membre ne compte plus de 3 000 habitants, d'une part, à déroger à l'interdiction de prise en charge, dans le budget général, des dépenses au titre des services publics, des services publics, d'autre part, à établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. Or ce seuil de population n'est aujourd'hui plus en phase avec la réalité de l'intercommunalité. Le ministère de l'intérieur en est d'ailleurs convenu dans la réponse qu'il a apportée, le 29 mars dernier, à la question écrite sur l'eau et l'assainissement n° 03368 de notre collègue Sophie Joissains. précisé qu'« une adaptation des seuils de population permettant d'établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement pourrait être étudiée

pour permettre la création d'EPCI dont la population est inférieure au seuil minimal, fixé à 15 000 habitants. Les EPCI concernés correspondent à des territoires ruraux et de montagne, pour lesquels ces exceptions à la prise en charge de dépenses du budget de l'eau par le budget général et à la tenue de deux budgets distincts pour l'eau et l'assainissement constituent des facilités essentielles pour la gestion par ces collectivités des services de l'eau et de l'assainissement. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par Mmes M. Carrère, Dans le même esprit, il s'agit de reprendre un article inséré dans la proposition de loi adoptée en février 2017 dans ce même hémicycle. Les articles L. 2224-1 et suivants du prévoient actuellement le principe de l'équilibre budgétaire des services publics industriels et commerciaux. À cet égard, les services publics de l'eau et de l'assainissement, qui sont des SPIC, y sont soumis. Le législateur a néanmoins introduit une dérogation pour les communes de moins de 3 000 habitants et les EPCI dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants. La nouvelle carte intercommunale vient bouleverser ces équilibres. Avec la fusion d'intercommunalités, ces dernières devront, lors de la prise des compétences « eau » et « assainissement », équilibrer leurs budgets annexes de l'eau et de l'assainissement par les seules redevances des usagers. Afin d'éviter une augmentation excessive du prix de l'eau et de l'assainissement pour les usagers lors du transfert de la compétence à l'EPCI, il est proposé de relever le seuil de 3 000 à 5 000 habitants pour les communes et les EPCI. permettra aux communes appartenant à une intercommunalité ne disposant pas de communes de grande taille de ne pas être pénalisées pour le versement de l'attribution de compensation quand leurs budgets annexes ne sont pas équilibrés. Par ailleurs, elle permettra aux EPCI au périmètre élargi de continuer de bénéficier de cette dérogation.

de la commission ? Les amendements n 24 rectifié et 9 rectifié ont pour objet d'élargir le champ de la dérogation permettant aux communes de verser une subvention d'équilibre au budget de leurs services de distribution d'eau et d'assainissement, et ce quel que soit leur mode de gestion. L'article L. 2224-2 interdit en effet par principe aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics à caractère industriel ou commercial. Il prévoit néanmoins, entre autres, une dérogation pour les communes de moins de 3 000 habitants et les intercommunalités ne comprenant aucune commune membre de plus de 3 000 habitants, pour ce qui concerne leurs services de distribution d'eau et d'assainissement. L'amendement n° 24 rectifié tend à supprimer ce seuil de population. L'amendement n° 9 rectifié a quant à lui pour objet de le relever à 5 000 habitants, compte tenu de l'élargissement des périmètres intercommunaux.

budget unique. En outre, le présent amendement est problématique sur le fond, dans la mesure où il conduirait à faire financer le coût du service par de la fiscalité,

des recettes au titre des redevances d'occupation du domaine public. Aujourd'hui, il semblerait que ces recettes soient transférées automatiquement aux EPCI.

alors que, à une certaine échéance, le transfert de compétences serait obligatoire. On peut imaginer que certaines communes feraient des travaux importants avant de transférer des soldes négatifs. Nous nous trouvons dans une situation de fragilité juridique très préoccupante.

Je rappelle que ces compétences relèvent d'un SPIC au travers des budgets annexes distincts du budget principal. À l'issue de l'étape budgétaire du transfert des compétences « eau » et « assainissement », les résultats budgétaires ou excédents de clôture du budget annexe communal, ainsi que les restes à réaliser sont nécessairement intégrés en totalité au budget principal de la commune. Autrement dit, les résultats budgétaires de l'exercice précédant le transfert de compétences sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils résultent de l'activité de celle-ci lorsqu'elle était compétente. Cela s'explique par le fait que les SPIC sont soumis au principe de l'équilibre financier qui nécessite l'individualisation des dépenses et des recettes au sein d'un budget spécifique, assortie de l'impossibilité de financement par le budget principal. De ce fait, les déficits et les excédents qui résultent strictement de l'exercice de la compétence peuvent être identifiés. Toutefois, pour les SPIC uniquement, les résultats budgétaires du budget annexe communal, qu'il s'agisse d'excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou partie. Ce transfert doit donner lieu à des délibérations concordantes de l'EPCI ou de la commune concernée. En d'autres termes, le transfert des résultats budgétaires à l'EPCI bénéficiaire d'un transfert de compétences représentant un SPIC ne constitue donc pas

Or il nous apparaît qu'une telle dérogation serait contraire aux principes mêmes qui régissent aujourd'hui les SPIC. Nous n'y sommes pas favorables, car un tel dispositif introduirait une dérogation au droit général des SPIC, ce qui ajouterait une complexité peu justifiée. La commission

en précisant que « le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public

Mon collègue Jean-Pierre Sueur vient d'évoquer la question orale posée à l'Assemblée nationale cela peut sembler de bon sens, mais un peu étonnant dans un État de droit -que cette décision du Conseil d'État n'interdisait pas les accords au sein du bloc communal. Mais quelle fragilité juridique,

unitaires ou non unitaires, en tout cas. Nous considérons que la commission des lois a déjà amélioré la rédaction de l'article 2 en rétablissant la sécabilité entre l'assainissement et la gestion des eaux pluviales. Toutefois, nous voudrions aller un peu plus loin par souci de clarification, afin de ne pas laisser place à une quelconque interprétation. C'est pourquoi cet amendement vise à exclure explicitement la gestion des eaux pluviales de la compétence « assainissement » et à permettre aux communautés de l'exercer de manière facultative. Quel est l'avis de la commission ?

opter pour la sécabilité entre ces deux compétences en retenant le dispositif déjà adopté par le Sénat le 23 février 2017 à l'article 4 de la proposition de loi Bas-Retailleau, sur l'initiative de notre excellente collègue Françoise Gatel. Gatel. Fidèles à cette philosophie, nous préférons laisser le soin aux élus locaux de décider de la sécabilité là où elle est justifiée. En effet, dans certains territoires, une gestion commune de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales nous paraît pertinente, dans d'autres moins. C'est pourquoi la commission

Une telle modification ne permet pas d'apporter par la loi une clarification quant à l'échelon auquel doit être assurée la gestion des eaux pluviales urbaines. C'était au contraire le sens de la solution proposée par M. de Belenet,

objet est de maintenir l'eau et l'assainissement dans les compétences des communes de la métropole d'Aix-Marseille Provence sur la décision de ses entités déconcentrées, les conseils de territoire, à qui ces compétences auraient été déléguées. Néanmoins, d'une part, l'eau et l'assainissement l'eau et l'assainissement relèvent des compétences obligatoires des métropoles et, d'autre part, si la métropole d'Aix-Marseille Provence, en vertu des compétences qui lui sont spécifiques, peut déléguer ces matières aux conseils de territoire, c'est à l'exception des schémas d'ensemble d'assainissement et d'eau pluviale.

Estrosi Sassone. L'article 3 de cette proposition de loi vise à assouplir les règles de représentation-substitution des communes au sein des syndicats exerçant les compétences « eau » et « assainissement » et à permettre aux syndicats regroupant deux EPCI à fiscalité propre de bénéficier de ce dispositif. Le rapporteur a jugé cet assouplissement bienvenu, car il permet de préserver de nombreux syndicats existants et d'assurer la continuité des services rendus aux usagers.

» dont la conséquence était la dissolution des syndicats ne regroupant pas au moins trois EPCI. En effet, il convient de prévoir une telle modification pour les métropoles, donc de l'étendre à l'article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales. À défaut, certains syndicats mixtes regroupant en leur sein des communautés d'agglomération et des métropoles seraient fragilisés et devraient disparaître. Cet amendement vise donc à permettre aux communautés d'agglomération et aux métropoles de maintenir les syndicats mixtes compétents en matière d'eau et d'assainissement dont elles seraient conjointement membres.

Il est ici proposé de modifier les dispositions de représentation-substitution. Le mécanisme permet d'assurer la pérennité des syndicats mixtes qui comprennent, dans leur périmètre, des communes appartenant à au moins trois à fiscalité propre différents. Les EPCI concernés ont alors vocation à se substituer à leurs communes membres au sein du comité syndical. L'article 3 de la proposition de loi prévoit un assouplissement de

pas, mais vous demandez que la règle prévoyant le retrait des communes membres des syndicats comprenant dans leur périmètre moins de trois EPCI à fiscalité propre soit maintenue s'agissant des métropoles-

Sans surprise, à l'issue de cet après-midi de débat, notre groupe votera le texte tel qu'il est issu des travaux du Sénat.

les dates de 2018 et de 2020 nous apparaissaient totalement absurdes et irréalistes. Nous l'avons défendue

En même temps, donc, nous sommes très attachés aux progrès en matière d'intercommunalité. Nous pensons qu'il doit être possible d'aller vers plus d'efficacité et de mutualisation, en particulier au regard du prix de l'eau et de la

de s'organiser librement, pour la plus grande efficience de leurs services. L'examen d'un certain nombre d'amendements déposés sur ce texte montre que l'on veut aussi définir, par la loi, toute une série de relations entre les collectivités qui doivent normalement rester contractuelles.

vote. Notre groupe Les Républicains reste très cohérent. Lors de l'examen de la loi NOTRe, nous étions opposés à toutes les mesures réduisant l'autonomie des communes, notamment sur deux points de nouvelles compétences obligatoires, que nous refusions, et l'élection au niveau intercommunal des conseillers communautaires-

et si elle adoptait l'élection des conseillers communautaires au niveau intercommunal, cette décision était irréversible, puisqu'elle s'appuyait sur le principe constitutionnel de l'action directe des élus des collectivités qui lèvent l'impôt.

et la nature ne délimitent pas les mêmes périmètres : un bassin de vie n'est pas un bassin versant, ni aujourd'hui ni dans quelques années. Nous rétablissons donc ce caractère optionnel ; il appartiendra à la nouvelle majorité de l'Assemblée nationale de confirmer ou non cette liberté rendue aux communes non pas pour préserver des prérogatives, mais pour choisir sur chaque territoire le mode de gestion le plus adapté aux problématiques locales. La parole

les maires, notamment ceux des communes rurales sont des gens pragmatiques, sérieux, qui connaissent et gèrent avec beaucoup d'attention et d'application l'eau et l'assainissement. Laissons-leur la liberté de transférer ou non la compétence aux communautés de communes. Vous avez, madame la ministre, apporté une amélioration à la loi NOTRe avec la possibilité de décaler le transfert en 2026. Toutefois, je soutiens la proposition de la commission d'un transfert optionnel des compétences « eau » et « assainissement », sans date, comme cela a été voté en 2017 par le Sénat. Les maires sont des gens responsables, soucieux de leur commune : nous devons leur faire confiance. La parole est à M. Olivier Paccaud, pour explication de vote.

d'eau, d'assainissement, et qui, dans beaucoup d'endroits, le font quasi bénévolement, c'est-à-dire avec des indemnités pharaoniques de 200 euros ou 250 euros par mois. Ils sont disponibles, compétents, ils connaissent parfaitement, sans être sourciers, les détours et les contours de leurs réseaux. Et si, malheureusement, que ce soit en 2020 ou en 2026, leur syndicat disparaît, j'ai bien peur que l'enjeu dont nous parlait Mme Gourault, à savoir la bonne gestion, la maîtrise des coûts de fonctionnement, soit perdu de vue,

Mme la ministre, dans son propos introductif, a insisté sur le fait que de nombreuses intercommunalités avaient déjà franchi le pas du transfert de compétences. C'est exact. Mais elle a sous-entendu que c'est parce que la démarche était logique et que les réseaux seraient ainsi mieux gérés. Mais la vérité, en tout cas dans mon département de l'Oise, c'est que ceux qui ont franchi le pas n'avaient qu'une seule motivation : les

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable sur la nomination de M. François Jacq aux fonctions d'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (n° 388, trente : Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, portant sur le projet de programme de stabilité pour 2018-2022, en application de l'article 50-1 de la Constitution. Suite éventuelle de la proposition de loi,